La séance est reprise. Les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour vous ont été adressées par courriel et sont consultables sur le site du Sénat. Elles seront considérées comme adoptées en l'absence d'observations d'ici à la fin de la séance.- fin de la séance.- Suite de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles en France continentale et dans les outre-mer

Le déclassement social de la paysannerie n'est pas une vue de l'esprit. Aujourd'hui les retraites agricoles demeurent très faibles, en comparaison de celles des autres régimes. Cela a maintes fois été rappelé aujourd'hui, mais aussi lors de nombreux travaux ici, au Sénat, ou à l'Assemblée nationale. Comment peut-on laisser vivre les agriculteurs sous le seuil de pauvreté, alors qu'ils sont la richesse de nos territoires et de nos terroirs ? Comment peut-on prétendre qu'ils peuvent encore attendre, alors que l'urgence sociale est là, sous nos yeux ? Comment pouvez-vous leur dire qu'ils peuvent attendre 2020, alors que vous vous êtes empressés, lors de votre premier budget, de rendre 3 milliards d'euros aux ultra-riches de ce pays ? Vous n'êtes pas le gouvernement des riches, vous êtes le gouvernement des nantis ! Nous avons la possibilité de changer le quotidien des agriculteurs immédiatement, sans contradiction avec la future réforme des retraites. Nous avons la possibilité d'augmenter d'un peu plus de 100 euros par mois le pouvoir d'achat des 230 000 bénéficiaires actuels du dispositif. Mais pour des raisons obscures, vous refusez tout simplement cette avancée que de nombreux retraités attendent. Alors que la France vient de se voir une nouvelle fois reconnaître le titre de « championne de monde du reversement des dividendes aux actionnaires » par l'ONG OXFAM, et et que les « premiers de cordée français sont les champions toutes catégories de la spéculation financière », il ne serait donc pas possible de prélever le minimum indispensable à la vie digne de nos retraités de l'agriculture. Vous avez soulevé bien des arguments techniques contre ce texte, qui ont tous été contredits. Vous avez mis en avant la précipitation avec laquelle les parlementaires auraient agi. C'est oublier que cette proposition de loi est le fruit d'un travail de terrain, d'auditions multiples, du travail des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces propos sont l'illustration du mépris de l'exécutif à l'égard du Parlement. Recours systématique aux ordonnances, à la procédure accélérée, au vote bloqué, au temps programmé, à l'utilisation détournée des armes du parlementarisme ce n'est pas seulement l'opposition qui est muselée, mais tout le pouvoir législatif que l'on tente de bâillonner. Le pseudo-renforcement de l'efficacité du travail parlementaire et de la productivité législative, ce ne sont que des mots creux

Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ? » C'est là le message aussi affligeant que navrant et inacceptable que vous adressez, avec votre gouvernement, madame la ministre, aux agricultrices et agriculteurs retraités, qui n'en peuvent plus d'attendre et qui ont assez vu le soleil poudroyer et l'herbe verdoyer. C'est un véritable SOS qu'ils nous adressent et que nous devons entendre dans cet hémicycle. En France continentale et en outre-mer, les pensions de retraite agricoles sont parmi les plus petites pensions de toutes toutes les catégories socioprofessionnelles. En 2015, la moyenne était de 790 euros bruts par mois pour un ancien exploitant, certaines n'atteignant même pas 500 euros. Les fédérations départementales d'exploitants agricoles ont rempli leur office. Mes chers collègues, comme moi vous avez reçu des dizaines et des dizaines de courriers d'agriculteurs et d'agricultrices, accompagnés des justificatifs de la MSA, indiquant la pension de retraite qu'ils perçoivent. Et comme moi dans l'Aude, vous avez pu prendre connaissance de ces montants. Combien sont en dessous du seuil de pauvreté ? C'est intolérable ! Véritable serpent de mer, ce problème a assez duré. Il faut agir ici et maintenant. J'aimerais pouvoir dire « avant qu'il ne soit trop tard ». Mais, malheureusement pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, il est déjà trop tard. Madame la ministre, vous avez pleinement conscience des embouteillages que connaît notre calendrier parlementaire, avec tous les textes qui sont en attente d'examen. Nous ne pouvons attendre que soit discutée une future réforme des retraites. Comment pouvez-vous d'ailleurs invoquer cet argument pour reporter l'application de cette loi, alors que nous ne connaissons pas les contours de cette future réforme ? de belles paroles, qui consistent à nous dire que « c'est une bonne idée mais, promis, on le fera plus tard et dans le cadre d'une grande réforme ». Croyez-moi, ces trois ans et demi de mandat sénatorial m'ont bien fait comprendre qu'il ne faut pas remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même

de dire notre reconnaissance à celles et ceux qui produisent notre alimentation, de redonner dignité et fierté à l'ensemble de ces femmes et de ces hommes qui cultivent et entretiennent nos paysages. Le Président de la République nous a annoncé un monde nouveau. N'était-ce pas là l'occasion de passer des promesses aux réalités ? Certes, vous annoncez une réforme systémique des retraites, et le temps ne serait pas aux exceptions. Je comprends ces scrupules respectables, mais ce texte n'est pas en contradiction avec de tels principes. Il prévoit simplement une anticipation. Parce que la situation des retraités agricoles est extrêmement difficile

Gouverner, c'est renoncer, disent certains. Gouverner, c'est aussi choisir, diront d'autres. Le groupe Union Centriste choisit d'apporter une solidarité morale et matérielle au monde agricole.

Madame la ministre, quelle est votre vision de la démocratie ? On a bien compris que tout se décide dans ce microcosme parisien, loin des territoires. Cela nous touche et nous déçoit. Il vous faudra bien plus qu'un direct avec Jean-Pierre Pernaut pour vous réconcilier avec la ruralité et l'agriculture ! Aucun corps

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, les enfants et les petits-enfants d'agriculteurs parsèment cet hémicycle. Ils ont écouté ce que portent de juste et de digne revendication ces femmes et ces hommes du XXsiècle qui ont pris de la peine sans s'enrichir et qui aujourd'hui ne sont pas reconnus pour ce que la Nation leur doit. Ces agriculteurs retraités, en tout cas leurs représentants, sont là ce soir, avec nous, et je veux avec vous tous les saluer pour leur combat, leur opiniâtreté à se faire entendre et reconnaître. Madame la ministre, il ne faudra pas nous dire, comme ce fut le cas le 7 mars dernier, qu'il fallait le faire avant. Parce que cette question du progrès des retraites s'inscrit dans un long processus que la famille politique qui est la mienne a impulsé, sous la gouverne de Lionel Jospin et de François Hollande. Pourquoi les progrès réalisés de 1997 à 2002, et de 2012 à 2017, ne pourraient-ils pas être poursuivis avec le texte porté par André Chassaigne ? Comment comprendre les arguments que vous avez développés le 7 mars ? Vous nous aviez expliqué que vous souhaitiez que ce sujet soit intégré dans la réforme des retraites que vous projetez, réforme construite sur le principe annoncé par le Président de la République du « 1 euro de capitalisation pour 1 euro de revenu Que donneront les retraites des agriculteurs qui aspirent légitimement aux 85 % du SMIC avec la mise en oeuvre de ce principe ? Ce qu'elles donneront, c'est une régression Depuis quelque temps, à grand renfort d'assises, d'états généraux divers et variés, la Nation se porte, à juste titre, au chevet de son agriculture, de ses producteurs qui se voient dérober la juste valeur de leur travail. Plus de 160 suicides en 2016, des histoires familiales marquées tragiquement pour des générations, des vies vidées de sens et de toute espérance, des conditions de vie précaires et parfois, trop souvent, indignes d'un pays développé : cette situation est intenable et ne peut plus durer Avec mes collègues du groupe socialiste et républicain, je plaide pour que nous ouvrions de nouvelles perspectives aux actifs, et je suis convaincu que la revalorisation des retraites agricoles doit et peut en faire partie, en complément de la reconnaissance de la juste valeur du travail de production.

La dimension morale d'une telle posture serait proprement abjecte, et elle est inconcevable dans le cadre des valeurs de la République. Pour ce que la Nation leur doit, les plus modestes des retraités agricoles de France méritent autre chose

500 euros pour les femmes. Tout a été dit aussi sur les procédures que vous avez utilisées pour éviter que se tienne un véritable débat de fond sur ce sujet. Je voudrais, en tant que sénateur de la Dordogne, dire que ces femmes et ces hommes ont un visage. Nous les connaissons.

qui représentent des milliers de retraités agricoles-6 000 en Dordogne -, savent ce qu'il faudra faire demain. J'espère donc que le vote sera unanime, ce soir, sur les travées du Sénat.

Mon propos sera rapide et clair : le simple fait, madame la ministre, de reporter par une manipulation réglementaire cette possibilité d'augmentation démontre, à mon sens, le mépris que vous avez pour le peuple des travailleurs de la terre, peuple dont je fais partie puisque je suis paysan. Une seule question

En reportant à 2020 la revalorisation des retraites, en arguant de l'équité entre les assurés sociaux, vous ne prenez pas en compte la situation inégalitaire qui perdure depuis des décennies pour des femmes et des hommes dont les pensions de retraite sont parfois

Enfin, en utilisant la procédure du vote bloqué, vous donnez une bien piètre image du débat public et de l'outil parlementaire. À l'heure où la défiance de nos concitoyens envers le politique atteint son paroxysme, ces agissements ne font que conforter les Français dans ce sentiment. Vous devez aujourd'hui prendre vos responsabilités quant à vos agissements. Nous prenons acte de votre décision, ce soir, de maintenir cette procédure antidémocratique, mais il appartient dès lors au Gouvernement d'expliquer pourquoi il laisse mourir de faim des femmes et des hommes qui ont travaillé tant d'années nourrir les femmes et les hommes de notre pays. Je le dis ici avec la plus grande solennité, ce que vous faites ce soir, finalement, c'est utiliser cette proposition de loi sur les retraites agricoles pour faire la démonstration que vous ne céderez sur rien. Mais en ne cédant sur rien, vous ne ferez pas avancer la démocratie. En ne cédant sur rien, vous ne créerez certainement pas le « nouveau monde ». Vous ne donnerez pas, en tout cas, l'envie aux femmes et aux hommes de notre pays de croire en la politique pour les années et les décennies qui viennent.

Madame la ministre, en janvier dernier, nous avons voté ici au Sénat une proposition de loi portant création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes des pesticides, aux premiers rangs desquels se trouvent Vous aviez exprimé votre opposition à la création de ce fonds, qui était pourtant attendue par les victimes. Le motif que vous avez invoqué était qu'il fallait attendre,

à Mme la ministre. Mesdames, messieurs les sénateurs, l'article 1 de la proposition de loi vise à relever le niveau minimal de pension perçue par un chef d'exploitation pour une carrière complète. Le présent amendement tend à reporter de 2018 à 2020 l'entrée en vigueur de cette disposition. Comme vous le savez, un débat va s'engager sur la réforme systémique de nos régimes de retraite. Il s'agit d'une réforme de grande ampleur qui vise à mettre en oeuvre un système plus équitable. La question du niveau minimal de pension qui doit être versée à un retraité ayant travaillé toute sa vie sera l'un des enjeux importants du débat dans le cadre de la mise en oeuvre de système universel de retraite. Cette question concernera l'ensemble des assurés sociaux, quel que soit le secteur d'activité professionnelle.

sur votre amendement, qui est loin d'être anodin. Au-delà d'une apparence de changement de date, c'est bien évidemment le sens même de la proposition de loi que vous remettez en cause. en cause. Les choses sont assez claires sur ce point. Je voudrais dire que j'ai pris plaisir à travailler avec la

le texte n'était pas financé- j'y reviendrai, il l'est : 450 millions d'euros de recettes pour une dépense de 400 millions d'euros -et que la réforme était prématurée. Allez le dire

par les retraités agricoles et par les territoires ruraux dans leur ensemble. C'est pourquoi je rappelle que la commission des affaires sociales a émis un avis défavorable sur cet amendement. Le vote est

madame la ministre, mes chers collègues, cet article de la proposition de loi porte sur le financement de la remise à niveau des retraites versées par le régime agricole. Bien entendu, ce ne serait pas la première fois qu'une recette de caractère fiscal serait mobilisée pour financer un des pans de « l'effort social de la Nation », puisque le régime agricole fait déjà l'objet de maintes dispositions de cette nature. Pourquoi une taxe additionnelle sur les transactions financières ? Tout simplement parce que, depuis l'adoption de la loi de modernisation des activités financières il y a plus de vingt ans, vingt ans, les produits agricoles sont entrés dans le circuit infernal des marchés financiers de toute nature. Il existe des contrats à terme pour négocier le prix des matières premières agricoles, en France, en Europe, comme sur d'autres places boursières où l'on échange la production de pommes de terre, par exemple, avant que celles-ci n'aient commencé de fleurir, où l'on trafique le cours des produits de première transformation, où l'on décide, devant un écran, du prix que l'on paiera à un éleveur laitier ou à l'éleveur d'un troupeau de vaches allaitantes ... Sans compter, bien entendu, les opérations menées sur les marchés céréaliers ! Soyons réalistes ce qui désorganise les prix agricoles depuis plus de vingt ans et crée, par conséquent, une forte incertitude pour les exploitants en activité et met en question la régularité des ressources de la Mutualité sociale agricole, ce sont bien les transactions financières de caractère spéculatif. à taxation est donc non pas une idée saugrenue ou une illumination de quelque intellectuel marxiste ou d'un intellectuel qui serait ni de gauche ni de droite, ou de gauche et de droite, mais une simple question de logique : que l'argent que l'argent du travail aille au travail, alors que la spéculation n'est rien d'autre qu'une ponction indue sur le travail ! Ne l'oublions jamais : les premiers marchés financiers à produits dérivés ont porté sur des produits agricoles. Il s'agissait alors de blé, de maïs, de viande de boeuf ou de jus d'orange. Il est donc grand temps que la sphère spéculative, qui gage une partie de sa rentabilité sur le revenu des agriculteurs en activité, mette la main au portefeuille.

collègues, cet article se fonde sur la réalité vécue par nombre d'anciens chefs d'exploitation ultramarins qui, pour la plupart, ne remplissent pas les conditions d'obtention des dispositifs de solidarité,

En effet, en outre-mer, seuls 23 % des monopensionnés du régime des non-salariés agricoles disposent d'une carrière complète les anciens chefs d'exploitation ultramarins ont cotisé en moyenne 8,5 années de moins dans le régime que ceux de l'Hexagone. Aussi, l'article 3 permettra aux chefs d'exploitation ultramarins de bénéficier du minimum de retraite garanti à 75 % du SMIC, sans devoir justifier d'une durée minimale d'assurance dans le régime, à condition toutefois de justifier d'une carrière complète dans l'ensemble des régimes.

puisque les accords entre les partenaires sociaux locaux nécessaires pour étendre la couverture de retraite complémentaire n'ont été signés qu'en Guyane et en Martinique, excluant de fait les salariés agricoles des autres territoires ultramarins. L'article 4 vise ainsi à étendre la couverture complémentaire à l'ensemble des salariés agricoles de ces territoires. Il prévoit de donner dix-huit mois aux partenaires sociaux, à compter de la promulgation de la loi, pour négocier. Au-delà de ce délai, l'État pourra généraliser l'extension par voie réglementaire, afin de permettre à tous les salariés agricoles ultramarins d'être couverts par une complémentaire retraite. Le vote est

dans les outre-mer, il m'a demandé de le remplacer. Le titre I du texte que nous examinons vise à garantir un niveau minimum de pension à 85 % du SMIC et de nouvelles recettes pour le financement du régime des non-salariés agricoles.

Pourtant, une erreur s'est glissée dans l'intitulé de la proposition de loi, puisque, si ce texte ne devait concerner que la France continentale et les outre-mer, la Corse en serait exclue, la métropole étant composée de la France continentale et de la Corse.

réservé. Je vais mettre aux voix l'ensemble de la proposition de loi modifiée par l'amendement n° 3 du Gouvernement, comme ce dernier l'avait demandé le 7 mars dernier. Madame la ministre, confirmez-vous le champ de la demande de vote unique ?

Il serait possible de faire une simulation de calcul des cotisations sur les services rendus par ces agricultrices et agriculteurs qui n'ont jamais été rémunérés. Je ne remonterai pas jusqu'aux pertes des dernières guerres, mais nous pouvons trouver toutes sortes d'exemples de cette rémunération qui n'a jamais été donnée à ces agricultrices et agriculteurs. Les temps changent. où l'on s'apprête à débattre d'une loi portant sur l'équilibre entre les relations commerciales, l'alimentation et le revenu des agriculteurs, il ne faut pas oublier

sur lequel ils auraient pu cotiser, on parviendrait à une somme bien plus importante que celle qui vous est demandée aujourd'hui. Madame la ministre, soyez une vraie politique ! Nous vous soutenons et vous soutiendrons face à votre administration et à votre Premier ministre, et nous vous en remercions d'avance. Nous l'avons dit précédemment, cette proposition de loi est attendue, même si elle ne règle pas tout et qu'elle n'est pas l'alpha et l'oméga de la problématique des retraites dans le monde agricole. Cette proposition de loi a été conçue et travaillée par l'Association nationale des retraités agricoles de France comme une première marche à franchir, faire en sorte que les retraités agricoles, qui ont aujourd'hui les plus petites pensions et, par conséquent, vivent en dessous du seuil de pauvreté, retrouvent ce temps de dignité nécessaire

Aucun agriculteur aujourd'hui ne pourrait se satisfaire simplement de cette réévaluation à 85 % du SMIC, mais c'est une première chose à prendre, à acter, pour engager ensuite les discussions et les négociations à venir.

Vous le savez, il ne s'agira pas de reprendre simplement ce que vous avez balayé, piétiné, depuis le 7 mars dernier, pour faire réussir et approuver la réforme que vous proposerez en 2020. 2020. Ce soir, avant de passer au vote, il faut apporter une précision : ce n'est pas le Sénat qui empêchera que, demain, les plus petites pensions agricoles soient revalorisées dans notre pays, mais c'est bien le Gouvernement qui, par l'utilisation de cette procédure du vote bloqué, sera responsable demain matin devant les retraités agricoles de la pension qu'ils toucheront à la fin des mois à venir. C'est donc votre responsabilité. Bien évidemment, sans surprise, nous ne voterons pas cet amendement que vous nous proposez. Le reste vous appartient, vous en assumerez la responsabilité. Pour terminer, madame la ministre, je vous ai entendue le 7 mars

aucune traduction parce que, en réalité, le vrai problème, c'était de dire oui ou non aux revalorisations des pensions agricoles ! De cela, vous ne voulez pas ; de cela, vous vous expliquerez devant les retraités agricoles demain ! La parole est à M. Martin Lévrier,

désireuse de connaître les attentes de ces femmes et de ces hommes qui le composent, Mme la ministre a, comme elle s'y était engagée et comme vous le savez, rencontré, aux côtés du haut-commissaire à la réforme des retraites, l'ensemble des organisations agricoles. la ministre ! Les premiers concernés eux-mêmes ont compris l'enjeu et la cohérence de la démarche du Gouvernement alors que la majorité sénatoriale feint ici de ne pas l'entendre.

vous le voulez. Donc, la FNSEA estime que l'objectif de revalorisation des retraites est une urgence pour l'ensemble des retraités actuels et à venir. Mais, à l'inverse d'un grand nombre d'entre vous, la FNSEA a compris l'importance de patienter jusqu'en 2020 pour que les minima de pensions agricoles soient équivalents à ceux des autres régimes. n'est pas vrai ! La FNSEA a compris l'importance de patienter jusqu'en 2020 pour traiter le problème de manière pérenne.

Face à une telle posture, que je n'ose imaginer politicienne, vous ne laissez d'autre choix à la ministre en charge du dossier que d'utiliser l'article 44, alinéa 3, de la Constitution Il n'est ni logique ni raisonnable de statuer aujourd'hui et pour un seul corps professionnel sur des questions qui sont au coeur de la réforme des retraites. Le groupe La République En Marche se prononce donc pour le vote bloqué sur l'article 1.

Madame la ministre,

Je veux vous rappeler que, derrière les feuilles de calcul de Bercy, il y a des gens, des hommes, des femmes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté.

Nous allons évidemment rejeter votre amendement, madame la ministre, car, sur l'ensemble de ces travées, chacun a compris qu'il s'agissait en vérité, malgré tous les artifices que vous utilisez, d'un enterrement de première classe de la loi que nous proposons et qui était pourtant soutenue par tout le monde. Mais je veux ajouter que je suis extrêmement choqué par par le fait que, après l'ensemble des interventions qui se sont tenues sur toutes les travées, vous n'ayez même pas pris la peine de répondre à un seul des arguments développés. Vous avez expédié, en peut-être quinze secondes, votre réponse

du mépris que le Gouvernement a affiché pour ce texte depuis la discussion de mars dernier : mépris pour ce texte de loi, mépris pour les retraités agricoles et pour le monde agricole auquel ce texte tentait d'apporter une petite bouffée d'oxygène dans un monde- reconnaissez-le -bien difficile pour eux, mépris pour le Parlement. Le Gouvernement est en train de prendre d'une fâcheuse habitude. Hier soir, à l'Assemblée nationale, il a réussi le tour de force, sur les violences sexuelles- un texte qui aurait pourtant, là aussi, pu faire largement l'unanimité du Parlement -, de fédérer l'ensemble des groupes, à part celui de La République En Marche, qui a suivi sans discussion le Gouvernement.

c'est aussi un message d'espoir que nous envoyons au monde paysan. Nous ne les abandonnerons pas, nous ne céderons pas au subterfuge que vous utilisez ce soir. Il faut que le monde paysan le sache, des élus comme ceux du groupe CRCE continueront

ancien monde » n'est pas opposé au « nouveau monde » ; notre seul souci est de faire en sorte que les « derniers de cordée » du monde agricole puissent avoir un espoir pour la fin de leurs jours. Voilà la mission qui doit être la nôtre. Voilà le doute que, je l'espère, vous allez enfin partager en nous écoutant

Tout cela ne démontre qu'une seule chose, c'est que vous avez une obstination totalement jacobine. Malheureusement pour vous, la France, c'est 80 % de territoires ruraux

Que vais-je dire à mes compatriotes agriculteurs, qui se battent au quotidien contre des maladies phytosanitaires- la science n'a aujourd'hui aucune solution -, qui se lèvent tous les matins en regardant le ciel, redoutant cyclones, raz-de-marée ou inondations, qui sont de plus en plus fréquents- on connaît les conséquences du réchauffement de la planète ? Comment pourrais-je leur expliquer que cette France qui trouvera des centaines de millions d'euros pour organiser des jeux, les jeux Olympiques de 2024- manifestation que je défends et que j'apprécie

Je voudrais des réponses, madame la ministre, parce que, une fois dans mon avion, j'aurai honte à l'idée de les affronter.

afin de laisser aboutir le processus législatif ». Si, ça, ce n'est pas un soutien à la proposition de loi que je défends en tant que rapporteur, je n'y comprends plus rien ! C'est vrai, vous évoquiez plutôt

L'objectif de revalorisation des retraites à 85 % du SMIC est une urgence pour l'ensemble des retraités actuels et à venir de la métropole et d'outre-mer » ; voilà ce que dit la FNSEA

Monsieur le président, monsieur le président de la commission des affaires sociales, monsieur le rapporteur, mesdames, messieurs les sénateurs, alors que vous vous apprêtez à voter, je souhaite répondre à vos interventions et même à vos interpellations. Vous avez beaucoup parlé de mépris

J'en retiens une évidence, partagée par toutes les organisations : l'insatisfaction des exploitants agricoles à l'égard de leur régime de retraite et leur souhait de le voir évoluer,

il faut de la lisibilité et de l'équité. Toutes les organisations considèrent que le régime des pensions agricoles est illisible à force de complexité, et que beaucoup de règles sont injustes et insatisfaisantes.

plus largement, c'est la prise en compte de la variabilité des revenus agricoles dans la constitution des droits à la retraite qui est l'enjeu de fond. Ces organisations ont également évoqué les différences avec les autres groupes professionnels dans les règles applicables au régime de pensions. De nombreuses questions ont été soulevées à ce sujet ; je veux citer en particulier les règles de cumul entre emploi et retraite, mais aussi les conditions de calcul des pensions de réversion et la situation des conjoints et des aidants familiaux. Lisibilité et équité, voilà ce que demandent les organisations agricoles ; lisibilité et équité, c'est aussi ce que propose le Gouvernement comme principes de construction de la réforme systémique des retraites. Le haut-commissaire et moi-même, répondant à l'invitation de la Haute Assemblée et de son président, avons eu l'honneur de lancer officiellement cette réforme le 16 avril dernier et d'engager les concertations. Celles-ci aborderont en particulier la place des mécanismes de solidarité, puisque c'est de cela que nous parlons, dans la constitution des droits à la retraite, mécanismes qui intéressent tant les exploitants agricoles que l'ensemble de nos concitoyens.

il a semblé au Gouvernement légitime de proposer, dans l'urgence, deux améliorations au régime des retraites à destination des exploitants agricoles contraints de quitter leur activité pour cause d'inaptitude

Il va de soi que cette proposition emporte un engagement formel du Gouvernement pour faire aboutir ses propositions. Je rappelle d'ailleurs que, malgré le vote unanime dont vous parlez, le gouvernement précédent n'était pas favorable à cette réforme.

! Une réforme d'ensemble est engagée, avec un calendrier très précis, puisque les concertations s'achèveront avant la fin de l'année

un seul corps professionnel sur les questions essentielles, notamment de solidarité, qui sont au coeur de la réforme à venir. Vous n'avez

mais surtout pour alerter l'opinion sur les graves dérives en cours, qui mettent en péril l'équilibre démocratique de nos institutions. Cette question n'est pas réservée à quelques spécialistes. Elle concerne intimement chaque citoyen.

du « vote bloqué » par le Gouvernement à l'encontre d'une initiative parlementaire, met en exergue la pression de plus en plus forte exercée par le pouvoir exécutif sur les assemblées, y compris dans le cadre de leur compétence historique d'élaboration de la loi. Ce qui a expliqué la forte réaction à ce coup de force, madame la garde des sceaux, c'est la prise de conscience que vous approchiez d'une ligne rouge au-delà de laquelle la Constitution au sens historique du terme, c'est-à-dire la République, fondée sur le respect de la séparation des pouvoirs, ne serait plus respectée. Cette inquiétude des parlementaires a pris corps sur la quasi-totalité des travées de cette assemblée au fil des mois passés. Le discours du chef de l'État au mois de juillet dernier à Versailles, long et parfois tortueux, pour ne pas dire complexe, était transparent sur un point : l'ambition de réformer le Parlement. Pour Emmanuel Macron, le fil de ce projet est la recherche de l'efficacité. Pour d'autres, dont nous sommes, au travers de ce discours qui prend tout son sens aujourd'hui, c'est l'affaiblissement des assemblées qui est recherché, leur « mise sous tutelle », comme l'a exprimé le président du Sénat le 9 mai dernier. Le futur Président de la République, peu disert sur son programme durant la campagne électorale, a été clair sur un point : son nouveau monde ne pouvait supporter la supposée lenteur de la fabrication de la loi, pourtant chère à Mirabeau, et montrait clairement du doigt dans une attitude profondément démagogique le Parlement et les parlementaires comme des stigmates de cet ancien monde qu'il fallait s'empresser d'effacer. En vérité, vérité, la volonté est d'adapter les institutions des démocraties au rythme de la mondialisation libérale et de les y soumettre. Faut-il rappeler que, au-delà de l'annonce de la réduction du nombre de parlementaires- sur laquelle je reviendrai -, Emmanuel Macron avait même affiché l'idée de réduire le temps législatif du Parlement à trois mois Je pense que cet objectif est maintenu par le projet de loi constitutionnelle présenté la semaine dernière et par la volonté affichée par la majorité de l'Assemblée nationale. La question des droits du Parlement, ce n'est pas la défense des intérêts de quelques notables. Défendre ses droits, ce n'est pas se satisfaire de l'État existant, c'est-à-dire d'assemblées déjà affaiblies, peu représentatives et n'ayant apporté aucune solution satisfaisante aux yeux d'une large majorité de nos concitoyens.

Ces attentes d'un mieux vivre, d'une vie sereine, loin des violences sociales et de la dureté de la vie quotidienne, les gouvernements et les majorités parlementaires successifs n'y ont pas répondu et ont souvent aggravé la situation. Emmanuel Macron a bien perçu cette profonde déception, cette grande attente, et il les utilise pour renforcer son pouvoir présidentiel, symbole d'une nouvelle pratique, en réduisant le pouvoir parlementaire, survivance pour lui des institutions de l'ancien monde. Le projet constitutionnel qui doit être examiné par l'Assemblée nationale pendant les vacances, alors que ce débat devrait avoir lieu au grand jour, confirme pleinement nos craintes. Il s'agit là, comme je l'ai dit dans le débat précédent, d'un élément clé du dispositif mis en place avec les projets de loi organique et ordinaire à venir visant à réduire la place du Parlement dans l'architecture institutionnelle de notre pays. Le droit d'amendement est clairement dans le collimateur du pouvoir exécutif. La limitation du débat aux seuls amendements ayant un lien avec le texte dès la première lecture est un moyen de tuer l'échange démocratique en annihilant l'initiative parlementaire. Depuis des années, mes chers collègues, nous alertons sur la limitation progressive du droit d'amendement. Combien de fois avons-nous indiqué qu'en acceptant telle ou telle restriction- par exemple, la règle de l'entonnoir, qui bride le dépôt d'amendements en seconde lecture, ou l'interprétation extensive de l'article 40 de la Constitution, qui supprime toute possibilité de proposition en matière budgétaire, le développement des irrecevabilités allant jusqu'à mettre en cause la possibilité pour le parlementaire de proposer la remise d'un rapport sur tel ou tel sujet tel ou tel sujet -, c'est l'affaiblissement progressif du Parlement qui était validé ? Cette obsession du tri entre bons et mauvais amendements, entre amendements justifiés ou pas, a peu à peu créé les conditions aujourd'hui d'un véritable assaut contre ce qu'il reste du droit d'amendement. Cette obsession de la rationalisation du travail parlementaire nous a amenés à la situation actuelle : des débats sans saveur, sans enjeu, sans confrontation d'idées ou bien peu, sans possibilité de véritables échanges sur des propositions alternatives. En quoi les débats approfondis d'hier ont-ils posé un problème démocratique ? Prenons le cas de la crise actuelle de la SNCF, dont le Gouvernement porte l'essentiel de la responsabilité. Au-delà des options de fond, le choix d'une méthode autoritaire, archaïque par sa violence, n'aurait-il pu être évité par un véritable débat au sein de l'entreprise elle-même pour commencer, et au Parlement ensuite ? Prendre le temps du débat n'est pas seulement un artifice démocratique. Cela permet aussi à la société de s'exprimer, de faire valoir ses inquiétudes, ses colères Si la parole est restreinte au Parlement, si le droit de proposition est éteint, il ne faudra pas s'étonner que le peuple trouve tout à fait légitimement d'autres voies pour s'exprimer. L'exercice de la démocratie en France ne peut être réduit à la seule utilisation du bulletin de vote hors de l'élection présidentielle, les élections législatives étant devenues devenues une sorte de vote complémentaire à l'élection du chef de l'État du fait de l'inversion du calendrier. Permettez-moi de m'arrêter sur cette question, car le temps me manquera. Restaurer la plénitude des pouvoirs du Parlement passe bien entendu par une modification du calendrier électoral pour revenir à des élections législatives qui précèdent l'élection présidentielle. Il faut changer de régime ! Cela passe également, nous y reviendrons dans le cadre du débat constitutionnel, par une restriction des compétences du chef de l'État, son mode d'élection devant être La question d'une meilleure représentativité des parlementaires est également posée. Et ce ne sont pas quelques gouttes de proportionnelle invalidées par le seuil de 5 % des voix permettant d'accéder à la répartition de trois sièges qui changeront la donne Pour en revenir à la question précise des prérogatives parlementaires, le temps du débat, le droit d'amendement, le temps de parole doivent d'être défendus avec acharnement pour ne pas définitivement accepter le transfert du pouvoir législatif au Gouvernement et à la présidence de la République. La remise en cause de la navette par le projet de loi constitutionnelle s'inscrit dans le même objectif. Au-delà de la question des bienfaits ou non du bicamérisme et des qualités ou des défauts du Sénat, il est clair que l'objectif est de faire basculer tous les restes du pouvoir législatif vers l'Assemblée nationale, soumise, comme je viens de l'indiquer, au pouvoir présidentiel par la nature même de son élection. Pour conclure le tout, Emmanuel Macron a décidé de liquider l'initiative parlementaire en accordant une nouvelle priorité pour l'examen des projets gouvernementaux, empiétant sur les temps réservés aux assemblées. Comme vous le constatez, mes chers collègues, l'addition est lourde. Je l'ai dit, les origines de ce coup de force remontent à loin, et il est impératif aujourd'hui de remettre à plat ce que doit être la place du Parlement dans nos institutions et, par là même, ce que doivent être les prérogatives des assemblées dans ce cadre. Cette réforme ne peut être parcellaire. Elle remet en cause l'organisation même de nos institutions. Nous aurons l'occasion dans les semaines à venir de mettre en avant nos propositions pour une nouvelle Constitution qui tourne le dos à la dérive autoritaire à laquelle nous assistons et qui redonne toute sa place au peuple, à son intervention. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous assistons à un coup de force qui est l'aboutissement d'un long processus. Comment ne pas évoquer, par exemple, l'abandon du pouvoir budgétaire aux autorités européennes par le biais du traité budgétaire européen ? Ce fut un coup important porté aux pouvoirs du parlement national. Le coup de force entamé dès l'été dernier avec le recours aux ordonnances pour casser le code du travail s'est poursuivi avec l'application de la loi sur la sélection à l'université avant même son examen par le Sénat. Le Gouvernement méprise le Parlement en considérant tout texte déposé comme adopté et passe à l'étape suivante. Ce mépris et ces coups de force à répétition exigent une prise de conscience, une réaction démocratique et républicaine forte. C'est pour cela que nous avons demandé ce débat et que nous nous opposerons avec force dans le rassemblement le plus large aux réformes profondément antidémocratiques annoncées ces derniers jours. La parole

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous débattons aujourd'hui de l'évolution du rôle du Parlement face au pouvoir exécutif. Il ne pourrait être de débat

remontons quelques instants, si vous le voulez bien, à la genèse de la V République. Les pères fondateurs souhaitaient rompre avec l'instabilité ministérielle caractéristique de la IV République en instituant un parlementarisme que l'on disait déjà rationalisé. Dans ce cadre, l'opposition parlementaire pouvait difficilement se faire entendre, et les possibilités pour l'Assemblée nationale de renverser le Gouvernement étaient limitées. La fonction de contrôle de l'action gouvernementale était en quelque sorte neutralisée, privant en partie le Parlement de son rôle de contre-pouvoir. L'affirmation de l'exécutif était au coeur du projet constitutionnel, volonté intimement liée à une vision dépréciée du pouvoir législatif, qu'il s'agissait de limiter. La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, marqua un tournant fondamental dans l'histoire de nos institutions. Après plusieurs décennies de subordination, les pouvoirs du Parlement ont été fort opportunément reconsidérés et la tutelle de l'exécutif singulièrement diminuée. le Gouvernement ne peut plus recourir de manière parfois abusive ou illimitée à l'article 49.3. Par ailleurs- c'est extrêmement important -, il n'est plus l'unique maître de l'ordre du jour, celui-ci étant partagé. Enfin, les droits de l'opposition ont été renforcés et propositions de loi améliorées par la réhabilitation des commissions, le débat parlementaire ayant aujourd'hui lieu non pas sur le texte proposé par le Gouvernement, mais sur un texte élaboré, et souvent amélioré,

qui ressemblent fort à une limitation des droits du Parlement. Sous couvert d'un souci d'efficacité, l'ordre du jour pourrait être confisqué aisément par l'exécutif. Dès lors qu'un texte relatif à la politique économique, sociale ou environnementale serait jugé urgent, le Gouvernement pourrait décider de l'inscrire en priorité à l'ordre du jour. Il y a un risque risque que les urgences se transforment en ordinaire et deviennent la norme, l'ordre du jour réservé aux parlementaires se réduisant comme peau de chagrin. Autre signe inquiétant : le Gouvernement envisage un droit d'amendement encadré par de nouveaux critères de recevabilité particulièrement sévères qui contreviennent au pouvoir d'initiative et à la liberté des parlementaires, alors que les textes adoptés par le Parlement sont aujourd'hui majoritairement des projets de loi et que l'amendement constitue notre principale arme législative- au sens positif et pacifique du terme. Enfin, le rôle de contrôle du Parlement sur l'action du Gouvernement est passé sous silence. C'est le grand oublié de la révision constitutionnelle, alors qu'il s'agit d'une mission essentielle Dans toutes les grandes démocraties libérales, les parlementaires devraient ainsi disposer de moyens d'action renforcés pour évaluer les politiques publiques et l'efficience de l'action publique. Disons-le clairement, le le travail parlementaire est perfectible ; il doit être amélioré et sans doute nous arrive-t-il souvent- il faut le confesser pour parler vrai et juste -de nous sentir encombrés

d'amendements, la responsabilité de l'exécutif ne doit pas être niée, car nous avons affaire à des projets de loi confus, insuffisamment préparés, voire fourre-tout

Gouvernement. La discussion parlementaire peut effectivement gagner en efficacité et en fluidité- le Sénat a d'ailleurs montré l'exemple. Nos deux assemblées ont tout à gagner d'une amélioration de la fabrique de la loi. Toutefois, les mesures envisagées ressemblent fort à une rationalisation aveugle du travail parlementaire et écornent sérieusement la capacité à agir du Parlement. Le Parlement- je pense que vous en serez d'accord, madame la garde des sceaux et ne doit pas être une chambre d'enregistrement ou d'exécution obligée des souhaits d'un gouvernement aussi légitime soit-il. La démocratie ne peut vivre que sur les deux piliers que doivent être un exécutif fort et un législatif fort. Toute réflexion sur l'évolution des droits du Parlement serait incomplète sans citer la fonction essentielle du Sénat qu'est la double représentation de la population et des territoires. Notre pays puise son équilibre et sa cohésion démocratique dans la diversité de ses deux chambres. Or la singularité du Sénat, chambre de la sagesse et de la réflexion, moins soumise à une opinion publique trop souvent volatile que l'Assemblée nationale, court le risque d'être dénaturée, puisque le Gouvernement entend limiter la navette parlementaire au détriment de la Haute Assemblée. Le texte prévoit que, en cas de désaccord entre le Sénat et l'Assemblée nationale et d'échec de la commission mixte paritaire à adopter une version commune d'un texte de loi, le Gouvernement pourrait demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement, privant le Sénat de son droit d'expression. Madame la garde des sceaux, c'est vraiment un sérieux et très mauvais coup porté au bicamérisme et à ce qui fait son intérêt, à savoir le dialogue et l'échange constructifs entre les deux chambres, qui donnent le temps nécessaire nécessaire à l'élaboration d'un texte plus juste, plus pertinent, comportant moins d'erreurs et de lacunes. Enfin, le bicamérisme peut constituer- je le dis avec beaucoup de gravité -un obstacle à l'omnipotence et à l'impétuosité d'une chambre unique mue par des initiatives trop souvent impulsives, depuis l'introduction du quinquennat, qui engendre trop souvent une soumission de fait de l'Assemblée nationale au pouvoir exécutif. Le Gouvernement veut réformer et réformer vite. J'aurais préféré qu'il veuille réformer bien. Cette impatience réformatrice fait fi du temps nécessaire et incompressible à la fabrication de la loi et au contrôle de l'exécutif. La démocratie a besoin de ce double

demain, ce qu'il sera et ce que l'exécutif fera des libertés et de l'autorité qu'il entend aujourd'hui requérir de nous, parlementaires ? Nous veillerons à ce que la Constitution protège la démocratie

Nul n'ignore dans cette assemblée le contexte historique qui a présidé à la naissance de la V République il y a maintenant soixante ans. L'instabilité gouvernementale de la III et de la IV

En synthétisant, on peut dire que notre Constitution a complètement déplacé le centre décisionnel de l'État, du Parlement vers l'exécutif. En clair, entre les élections en France, c'est à l'exécutif qu'il revenait de déterminer les orientations de l'action politique.

la fonction présidentielle. Cette dernière concentre tous les pouvoirs- hors cohabitation -et les conserve, du moins dans leur faculté d'empêcher, pendant cette cohabitation. Par ailleurs, on le sait, le passage au quinquennat le passage au quinquennat et l'organisation des élections législatives à l'issue de l'élection présidentielle rendent désormais presque improbables les périodes de cohabitation, les élections législatives faisant office de lune de miel dans la mesure où elles ne sont que des élections de confirmation. Du point de vue symbolique, le fait que le Président de la République apparaisse dès le titre II de notre Constitution est sans doute révélateur. Je ne vais pas citer l'ensemble des articles qui montrent sa puissance, mais je rappelle que

Compte tenu de l'accumulation de toutes ces dispositions, les experts sont unanimes pour classer notre parlement parmi les parlements faibles au niveau international. Je tiens à préciser que, même après la réforme de 2008,

Les réformes successives ont tenté de corriger cette tendance inhérente à la V République. Je tiens cependant à souligner qu'elles ont toutes été menées dans le sens de nouvelles conquêtes pour le Parlement et que, la plupart du temps, on a fait appel à des comités d'experts, qu'ils soient présidés par des élus ou par des universitaires, pour tenter de corriger les maux connus de notre Constitution.

de 1958, à une période où le Parlement était infantilisé. Dans sa récente adresse au Parlement européen, le Président de la République a appelé l'Europe à résister aux tentations autoritaires. Heureuse inspiration sémantique quand le projet de réforme institutionnelle qui nous est présenté revêt précisément toutes les caractéristiques de l'autoritarisme

le Gouvernement nous propose tout simplement d'y mettre fin en empiétant sur l'initiative parlementaire et, par conséquent, en réduisant les droits des groupes minoritaires et d'opposition. Le Sénat a su faire preuve de sérieux pour limiter l'inflation du nombre d'amendements, mais ce n'est manifestement pas suffisant. Au lieu de s'interroger sur la qualité initiale de la loi, des études d'impact ou la nature fourre-tout de certains textes, le Gouvernement renforce ou veut renforcer les irrecevabilités pour encadrer au maximum le droit d'amendement, qui est essentiel à la fabrique d'une loi

Que dire encore de la réforme de la navette parlementaire, qui réduit tout simplement le Sénat à un rôle de spectateur, alors que sa mission est essentielle au fonctionnement du bicamérisme ? Il n'y a aucune efficacité à la dégradation du travail parlementaire, à plus forte raison quand il s'agit de la loi de finances, poussant ainsi subtilement à adopter le budget par ordonnances. Je vous le rappelle, l'Allemagne adopte ses textes en moyenne en 152 jours, contre 149

du renouvellement complet du Sénat en 2021 qui nous est proposé, la dernière surprise ? Alors que le renouvellement partiel du Sénat, chambre de la continuité, est une garantie de la stabilité des institutions, le Gouvernement innove en proposant la dissolution de la chambre haute

En usant à l'envi de la sémantique managériale, le Gouvernement ne pose pas les bonnes questions et apporte donc de mauvaises réponses. Car la première question que nous devrions nous poser est la suivante : si chacun s'accorde à dire que la fabrique de la loi peut être améliorée, que la démocratie doit être revitalisée, sur quel diagnostic se fonde cette réforme ? Quel est le sens de cette réforme ? Apporte-t-elle des réponses au désenchantement démocratique ? Remet-elle le citoyen au centre de la décision ? Que nenni ! En définitive, cette révision constitutionnelle semble être celle de l'exécutif pour l'exécutif et par l'exécutif : elle incarne l'hyperconcentration des pouvoirs, la crainte d'un débat parlementaire contradictoire, qui est l'essence de la démocratie, et l'éloignement démocratique.

De ce point de vue, la proposition qui nous est faite va vers une impasse démocratique ; elle ne mesure à aucun moment le danger que représente une telle atrophie dans le temps des contre-pouvoirs. Pour ces raisons, l'ensemble du groupe socialiste s'est

du général de Gaulle en 1946 : « Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : " Quelle est la meilleure Constitution ? " » Il répondait : « Dites-moi, d'abord, pour quel peuple et à quelle époque ? »

Que cette parole forte, qui a inspiré la V République, puisse nous porter et qu'elle fasse revenir le Gouvernement sur sa volonté actuelle de bâillonner le Parlement !

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, en 1958, afin de mettre fin à des années d'instabilité gouvernementale ayant marqué la fin de la IV République, les rédacteurs de la Constitution ont multiplié les instruments donnés au Gouvernement pour assurer sa stabilité et ses moyens d'action. Ainsi, le Parlement s'est vu, dès la naissance de la VRépublique, limité dans sa fonction législative. L'un des objectifs affichés de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a nécessité la modification de plus de la moitié des articles de la Constitution, a été de renforcer le Parlement législateur, en passant tout à la fois par une réappropriation de la procédure législative par les deux assemblées et une revalorisation de la norme législative. Si un certain nombre de dispositions ne concernaient pas directement le Parlement, en revanche, l'essentiel de la révision tendait à établir un nouvel équilibre entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. La réforme constitutionnelle de 2008 a ainsi permis de revenir sur des éléments souvent considérés comme fondateurs de la V République, tels que l'impossibilité pour le Président de la République de s'exprimer lui-même devant le Parlement, l'interdiction faite aux assemblées de voter des résolutions à l'adresse du Gouvernement, la prédominance du Gouvernement sur l'ordre du jour des assemblées ou encore l'engagement de la discussion législative sur le texte du Gouvernement et non sur celui de la commission. La révision de 2008 est à l'origine d'évolutions majeures : un nouveau partage de l'ordre du jour, le renforcement du rôle législatif des commissions, l'instauration d'un délai d'examen des textes, de nouvelles règles de présentation des projets de loi, la précision des règles de recevabilité des amendements, de nouvelles prérogatives pour les présidents d'assemblée dans la procédure législative, un encadrement du recours à l'article 49.3, la reconnaissance de droits aux groupes d'opposition ou minoritaires ou encore le développement du rôle du Parlement en matière internationale et européenne- tout en n'étant pas exhaustive, cette liste montre bien l'importance de cette révision. C'est non pas seulement le rôle législateur du Parlement qui a été renforcé à cette occasion, mais également le Parlement contrôleur. Néanmoins, je crois que nous pouvons admettre collectivement que nous ne nous sommes pas approprié l'ensemble des moyens constitutionnels à notre disposition pour ce qui concerne la fonction de contrôle. Avec Avec la révision qui s'annonce cette année, nous avons une occasion de conforter le travail de rééquilibrage des institutions commencé en 2008. La semaine dernière, vous avez présenté, madame la garde des sceaux, le projet de loi constitutionnelle pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace. Nous partageons avec le Gouvernement et le Président de la République ce triple objectif. Le texte présenté constitue l'aboutissement d'une annonce faite par le Président de la République à l'ensemble des parlementaires réunis en Congrès le 3 juillet 2017. Néanmoins, ce projet de loi constitutionnelle soulève plusieurs interrogations quant à l'équilibre nouveau trouvé en 2008. En premier lieu, le texte présenté le texte présenté envisage d'encadrer le droit d'amendement des parlementaires. La limitation d'un tel droit conduirait à un renforcement de la prédominance du pouvoir exécutif. Cela risque d'ailleurs de poser un problème constitutionnel, puisque le droit d'amendement est une liberté fondamentale des parlementaires qu'une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel a eu à coeur de garantir. Contraindre davantage cette liberté limiterait un droit consubstantiel au mandat parlementaire, qui est le sens même de la fonction de législateur, même s'il faut bien considérer que, parfois, des amendements présentés sont extrêmement éloignés des débats. Il est peut-être opportun de trouver des solutions à ce problème. En deuxième lieu, il est proposé de modifier le fonctionnement de la navette parlementaire. En cas de désaccord avec le Sénat, l'Assemblée nationale ne serait plus amenée à se prononcer sur la version sénatoriale. Évidemment, l'objectif final

de vouloir modifier le principe de l'ordre du jour partagé, en permettant au Gouvernement de le fixer prioritairement dans certains cas, cela ne peut se faire au détriment du rôle même des assemblées. Il y va du nécessaire équilibre institutionnel instauré par la réforme constitutionnelle de 2008. Cela conduirait à accorder au pouvoir exécutif une prérogative qui, à mon avis, prédominerait excessivement sur celle du Parlement. Madame la garde des sceaux, mes chers collègues, si la volonté du Gouvernement de vouloir répondre aux attentes de nos concitoyens en rationalisant davantage le fonctionnement du Parlement est louable et souhaitable, nous sommes tous attentifs sur les points que je viens d'aborder et qui ont été évoqués précédemment par d'autres orateurs, et des discussions seront nécessaires tout au long de la procédure parlementaire. y prendra pleinement part lors des prochains débats parlementaires, tout en restant ouvert à l'idée d'une plus grande célérité et d'une plus grande efficacité des travaux parlementaires. Exécutif et législatif ont tous deux le même objectif : la réussite de la France. La parole

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, la nature des relations entre le Parlement et le Gouvernement est un sujet de premier ordre dans une démocratie : elle mérite que l'on s'interroge plus encore à l'approche d'une importante réforme constitutionnelle. Depuis l'installation d'un régime parlementaire sous la III République, les droits du Parlement ont régulièrement évolué sous l'effet de révisions constitutionnelles, mais également en fonction de pratiques institutionnelles variables. Ils ne peuvent donc jamais être regardés comme acquis et doivent sans cesse être défendus par ceux qui ont reçu un mandat de la Nation et qui sont résolus à l'honorer. La défense de ces droits commence par leur exercice plein et entier le droit de questionner et de contrôler l'action gouvernementale, mais également le droit de proposer des textes de loi de leur propre initiative ou d'amender ceux qui sont soumis à leur examen. Plusieurs des grands progrès intervenus sous la IIIet la IV République sont à mettre au crédit de parlementaires, en particulier les radicaux, qui ont eu l'ambition d'exercer pleinement les droits attachés à leur mandat. Je pense en particulier aux lois scolaires soutenues au Parlement par les « Républicains opportunistes » et à la loi de séparation des Églises et de l'État, dont l'équilibre final fut imposé par la chambre des députés au ministre, conduite par son rapporteur Aristide Briand. Ironiquement, c'est pourtant le nom du ministre Émile Combes, le « petit père Combes », qui est resté pour la postérité Les fondateurs de la VRépublique, constatant les limites des précédents régimes liées à l'instabilité gouvernementale, ont considérablement encadré les droits des parlementaires, au nom d'un parlementarisme dit « rationalisé ». Le droit d'interpellation, redouté par tous les présidents du Conseil, qui étaient les Premiers ministres de l'époque, a été réduit à néant avec l'instauration de la procédure de motion de censure à l'article 49. Le droit d'amendement a également subi d'importantes limitations, en étant restreint au domaine de la loi, explicitement défini dans le texte constitutionnel, et considérablement encadré par la règle de l'irrecevabilité financière. Quant à l'initiative parlementaire des groupes minoritaires ou d'opposition, elle a disparu jusqu'à la révision constitutionnelle de 2008 et l'introduction d'un ordre du jour réservé. Mais, en parallèle, la croissance de la production normative européenne continue de représenter un défi pour notre parlement, qui reste relativement peu associé aux travaux des institutions européennes en comparaison des pratiques que l'on observe ailleurs, comme en Allemagne. Il faut y ajouter les les faibles pouvoirs de contrôle, alors que le champ et les moyens des commissions d'enquête sont considérablement encadrés par le droit et la jurisprudence constitutionnels, contrairement à ceux dont jouissent la Chambre des représentants et le Sénat américains. Pourtant, malgré sa capacité d'action contrainte, y compris après le rééquilibrage institutionnel de 2008, la Haute Assemblée a toujours fait un usage raisonné de ses droits : l'obstruction y est rare et le manquement aux règles des irrecevabilités y est strictement sanctionné. Lors de l'examen de la loi pour un État au service d'une société de confiance en commission, trente-cinq amendements ont ainsi été déclarés irrecevables au titre de l'article 45 et cinq au titre de l'article 40. La récente adoption de la procédure de législation en commission, la PLEC, illustre par ailleurs la capacité de notre institution à s'autoréguler, dans un souci d'efficacité législative. nous restons attachés à la conception du parlementarisme des jeunes radicaux que décrivait Jean Jaurès dans du 30 juillet 1887, c'est-à-dire une méthode de travail où des « efforts incessants de conciliation et de transaction permettent de dépasser les clivages et soutenir les progrès sociaux et économiques. Or cette conception implique de laisser les parlementaires exercer leur droit d'amendement dans des conditions symétriques à celles du Gouvernement. Nous considérons en outre que l'existence de discussions sincères et développées au Parlement est la meilleure réponse que nous puissions apporter au besoin de transparence de nos concitoyens, devenu impérieux. La publication des amendements soutenus par chaque parlementaire permet justement une grande traçabilité de l'activité des uns et des autres, donc de leurs responsabilités. De même, la publicité des débats permet également l'explicitation d'arbitrages réalisés au niveau interministériel et de s'assurer que l'ensemble des intérêts ont été pris en compte. Il n'est pas anodin que ce débat proposé par le groupe communiste se tienne dans le contexte particulier né de l'utilisation du vote bloqué sur une proposition de loi visant à revaloriser les pensions de retraite agricoles. Il intervient également après plusieurs réformes ayant contribué à affaiblir indirectement la capacité des parlementaires à apporter des solutions concrètes aux attentes de leurs concitoyens sur le terrain, qu'il s'agisse de l'encadrement du cumul des mandats ou de la suppression de la réserve parlementaire. En cherchant la vertu à tout prix, on crée des parlementaires hors sol. L'inadéquation entre les moyens juridiques accordés aux parlementaires et la grande responsabilité collective que leur attribuent les citoyens, par leur appartenance à ce qu'on appelle la « classe politique », a atteint sur ce sujet un point critique. Ce constat constituera le point de départ de la réflexion que le groupe du

Ces institutions, que d'aucuns voudraient bouleverser, ont évité à notre pays de connaître des crises politiques majeures, l'instabilité politique ou, comme nos amis italiens, la paralysie politique, source de fragilités dont l'histoire a pu nous apprendre qu'elles peuvent se révéler dramatiques dans certaines circonstances. Parmi les raisons essentielles qui fondent notre régime actuel figure la recherche d'un équilibre entre la légitimité présidentielle, voulue par son premier Président et destinée à doter les institutions d'un garant et d'un arbitre, et la légitimité des parlementaires, chargés d'écrire la loi et de contrôler l'action du Gouvernement. Ils sont nos blocs de marbre qui fondent nos institutions et qui ont pu admettre et supporter les nombreuses révisions de notre Constitution, et ce sans que soit remise en cause cette mécanique délicate construite autour de cet équilibre. révisions ont permis d'en peaufiner le fonctionnement et de l'adapter aux nouvelles réalités, notamment européennes. Mais elles ont surtout affiné le rôle du Parlement. Sans redevenir source d'instabilité politique comme sous la III et, plus encore, la IV République, elles ont renforcé ses moyens d'exercer au mieux son rôle d'artisan de la loi et de contrôleur de l'exécutif. Parmi celles-ci, la réforme de 1974 permettant à soixante sénateurs ou soixante députés de déférer une loi devant le Conseil constitutionnel ne fut pas la moindre. Depuis 1995, le Parlement siège en session unique ; depuis 2008, ses pouvoirs de contrôle ont été rénovés en profondeur et son fonctionnement a gagné en liberté et en modernité. Pour autant, il serait dommageable de rester béat : la V République souffre de maux qui lui sont propres, et ses institutions ont connu leur part de dérèglements. Songez donc au passage du mandat présidentiel

y a bel et bien des améliorations depuis le « parlementarisme rationalisé » des origines de la V République vers un « parlementarisme rationnel ». De son côté, l'actuel chef de l'État et l'exécutif laissent entendre que cette direction n'est pas la bonne. À ce stade, les annonces faites sur la prochaine réforme constitutionnelle semblent indiquer que l'exécutif serait insuffisamment doté des outils nécessaires pour gouverner. En tout cas, tel est le credo présidentiel. Qui peut croire sérieusement que la Constitution forgée par le général de Gaulle souffrirait presque d'un excès de parlementarisme ? Un argument massue est avancé : rendre le travail du Parlement plus efficace. « Plus, plus vite », nous dit-on. La commission mixte paritaire n'aboutit pas ? Eh bien, finissons-en au plus vite ! Le projet de loi de finances fait l'objet de discussions prolongées ? Une perte de temps inutile Cet amendement n'a qu'un lien indirect avec le texte discuté ? Il n'a pas lieu d'être ! Soyons francs, ce prurit réformateur ne me paraît pas compatible avec le coeur et l'essence même du travail parlementaire qui, par nature, demande du temps. En tout état de cause, il ne doit pas conduire à limiter la capacité du Parlement à remplir son rôle, celui que lui avait assigné le constituant, à savoir élaborer la loi et contrôler l'action du Gouvernement. Or, pour faire la loi, il faut certes de la rigueur, du dialogue, mais aussi, et surtout, du temps. L'un ne peut se faire sans l'autre. Nous avons tous des exemples de lois express, bâclées par une mauvaise impatience et tronquées par une précipitation. Songez que la loi de 1881 sur la liberté de la presse a été discutée devant le Parlement pendant près de six mois de 1905 de séparation des Églises et de l'État, devant laquelle notre collègue Requier a fait sa génuflexion, a fait l'objet de travaux et de débats durant près de neuf mois. Plus récemment, la loi Neuwirth légalisant la contraception a, quant à elle, été traitée pendant sept mois. Il est probable que le temps qui s'est révélé nécessaire à l'élaboration de ces lois ait fortement favorisé leur pérennité. Sur chacun de ces sujets, le temps consacré par le législateur aux débats n'a pas été perdu. Au contraire, il a été source d'enrichissement de ces textes, à la fois par des questionnements, des confrontations, des apports en termes de contenu et par l'onction mûrement réfléchie de la représentation nationale. Un autre aspect préoccupant de la réforme des institutions promise par l'exécutif est l'affaiblissement du Sénat. Notre « grand Conseil des communes de France », comme l'exprimait Gambetta, est trop souvent présenté comme un poids dans le processus législatif, voire un obstacle à la réalisation de l'intérêt général. Quoi qu'en dise, par lapsus ou non, le Gouvernement, madame la garde des sceaux, il y a un risque qui n'est pas fantasmé : le pouvoir exécutif, emporté en quelque sorte par l'présidentielle, à laquelle peut être soumise toute personne qui se sent consacrée, cherche à diminuer le rôle du Parlement Parlement par la réduction du droit d'amendement ou par la reprise en main de l'ordre du jour. Au bout du compte, le Gouvernement considère que cet espace commun consacré à la délibération que constitue le Parlement est un attribut superfétatoire ou un élément décoratif. Le temps nécessaire à la délibération est la condition de forme pour que le Parlement soit véritablement le lieu solennel et souverain dévolu à la fonction législative. « Les mots savent de nous des choses que nous ignorons d'eux », écrit le poète. C'est aussi vrai pour le débat parlementaire. En effet, la délibération permet souvent d'aboutir à une position ou à une analyse que l'on n'aurait pas eue tout seul ou que l'on n'avait pas eue initialement. Nous devons donc sanctuariser ce lieu. Le Sénat n'est certes pas un pouvoir d'opposition systématique, pas plus qu'un contre-pouvoir stérile : s'il peut être parfois un contrepoids, il est surtout un lieu de propositions et d'enrichissement de la loi. Madame la garde des sceaux, on n'a jamais vu un pouvoir périr de trop de débats. En revanche, on voit des pouvoirs s'atrophier en cédant à la tentation présidentielle du monologue, fût-il agrémenté et festonné des apparences du débat. Il est certain que la tentation présidentielle de décider seul est forte, mais c'est précisément notre rôle de mettre en garde contre ce prurit, qui ne peut qu'aboutir à une fausse réponse et, au final, à affaiblir la démocratie parlementaire- pléonasme précieux -, à laquelle nous tenons, madame la garde des sceaux.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, je souhaite tout d'abord saluer la démarche, à tous égards honorable, de nos collègues du groupe CRCE, qui nous convient à un travail d'examen critique de la pratique institutionnelle actuelle sur le point particulier, mais central, de la relation entre l'exécutif et le Parlement. Toutefois, je n'avais pas lu le sous-titre,

et, autant que possible, la rendre pertinente et, d'autre part, la capacité des deux à dialoguer lorsque le Parlement, au nom du peuple, exerce une fonction de contrôle.

? Concernant la contribution des deux composantes à la fabrication de la loi, j'observe dans tous les pays-

de loi, y compris dans les régimes facialement les plus parlementaires. Si vous prenez de temps en temps quelques minutes pour observer la vie politique et institutionnelle britannique, rien n'est plus évident. Il y aura toujours un équilibre ou plutôt en réalité- soyons francs entre nous -un déséquilibre entre l'initiative gouvernementale et l'initiative parlementaire pour l'engagement d'une proposition législative. En revanche, pour ce qui est du travail sur le projet, l'objet, la finalité sont, je le rappelle, une condition de la loyauté et de la transparence du débat parlementaire. Si l'objet même de la loi

donc cohérent et éthique du point de vue de la mission même du législateur de cadrer et de fixer les termes de l'objet législatif et du processus qu'il va traverser.

La Constitution prévoit déjà, sans que cela démange trop le Parlement depuis soixante ans, de ne pas présenter d'amendements sortant du domaine législatif, lequel est précisément encadré par la loi.

générale, le travail d'évaluation des commissions est très développé. Tout cela donne une production très riche. Simplement, comme le jeu ce soir semble être, pour le principal, de distribuer des mauvais points à l'exécutif, je voudrais que nous ayons un tout petit regard

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, lorsque, au groupe communiste républicain citoyen et écologiste, nous pensons à une réforme de la Constitution, nous avons tendance à l'envisager avec une visée l'émancipation humaine. Quand cette réforme touche aux institutions, au champ de la représentation, nous ne pouvons la concevoir sans l'idée d'introduire de nouveaux droits, tant pour les citoyens que pour le Parlement. Les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, qui composeront le projet de réforme des institutions ont récemment été transmis au Conseil d'État. en croire leurs intitulés, ils viseraient une « démocratie plus représentative et efficace ». Ils ne répondent pourtant ni à l'un ni à l'autre de ces objectifs. En vérité, cette proclamation n'est qu'une fable racontée par un système en crise. Cette crise est celle de la démocratie et de ses institutions. Jamais, en effet, une révision constitutionnelle n'est venue diminuer ainsi les pouvoirs du Parlement Baisse conséquente du nombre de parlementaires, attaque sournoise contre le droit d'amendement, dangereuse accélération de la procédure législative et de celle du vote du budget- laquelle

Montesquieu a dit : « Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. » Or s'il y a bien une chose que ces projets ne prévoient pas, ce sont des contre-pouvoirs. La réforme est une attaque portée au bicamérisme et à la démocratie parlementaire, parce qu'ils sont l'expression et le gage des contre-pouvoirs institutionnels. Car ce qui est mis en oeuvre, c'est un programme de renforcement pernicieux de l'exécutif et de disparition des idées différentes. Si le Parlement est la cible du Président, c'est justement parce qu'il est le lieu de représentation du peuple français et des territoires de notre pays, dans toute leur diversité. La défiance de l'exécutif à l'égard du pouvoir parlementaire traduit ainsi celle qu'il nourrit envers les citoyennes et les citoyens. La modification des modes de scrutin et la réduction du nombre des parlementaires vont non seulement éloigner le peuple de ses représentants, mais aussi renforcer davantage encore les logiques de polarisation et d'éviction des opinions situées aux extrémités du champ politique.

Que pèsent quelques dizaines de parlementaires ainsi élus face à l'amputation subie par des départements comme les Bouches-du-Rhône, la Seine-Maritime, le Nord, les Hauts-de-Seine, le Puy-de-Dôme ou encore la Seine-Saint-Denis, pour ne citer qu'eux, qui perdraient près de la moitié de leurs représentants Cette réforme promet de faire apparaître sur la carte de France de la représentation politique un monochrome inquiétant ! La réduction des pouvoirs du Parlement se fera au profit des technocrates, d'un gouvernement d'experts et de manageurs, qui, sous leur double casquette- certains sont experts et manageurs, suivant leur période de temps d'exercice professionnel -, croient croient détenir des vérités générales, considèrent les opinions divergentes et plurielles avec mépris, comme on l'a vu précédemment, et pensent qu'il n'existe pas plusieurs façons de voir le monde, mais seulement celle des détenteurs du pouvoir. Cette loi est un verrou elle ne vise qu'à tout clôturer, tout cloisonner, tout enfermer ! Il s'agit de museler les oppositions, les contestations, les propositions alternatives à celles que dicte la loi du marché. Elle est un outil au service de la stratégie managériale d'un Président qui considère la France comme sa start-up, exigeant sacrifices, obéissance et entrain pour la mise en place d'une politique qui ne sert que les intérêts privés des plus privilégiés. Rien ni personne ne doit être en mesure de proposer un autre horizon que la marchandisation du monde ! Or le Parlement n'est pas et ne doit pas se limiter à être une chambre d'enregistrement des décisions gouvernementales. Le Parlement est et doit être encore davantage une institution de contrôle du pouvoir, mais aussi une force de proposition de lois. Le Parlement est et se doit d'être toujours plus le témoin et le représentant de la diversité du peuple de notre pays. Madame la garde des sceaux, où sont l'audace et la modernité dont se targue pourtant si souvent le Gouvernement dans la réforme qu'il propose ? Une réforme constitutionnelle moderne et ambitieuse ne peut être qu'une réforme permettant l'éclosion de droits de droits nouveaux et progressistes, loin des logiques et des stratégies électoralistes visant à asseoir encore davantage le pouvoir en place, à délégitimer l'opposition et à faire taire toutes les formes de contestation. Une réforme constitutionnelle moderne et ambitieuse est celle qui traduit la confiance dans la démocratie et le Parlement, par exemple en inversant le calendrier des élections. Mettez les législatives avant la présidentielle ! Ce Elle est aussi celle qui parvient à traduire le pluralisme social en un principe de fonctionnement de nos institutions. Une réforme constitutionnelle moderne et ambitieuse doit ainsi être celle qui ancre dans ses gènes le droit de vote des étrangers et le principe de solidarité qui doit unir la fraternité humaine. Une réforme constitutionnelle moderne et ambitieuse doit avoir à coeur de penser toutes les procédures et tous les rouages inhérents à l'organisation du système démocratique, autour d'un impératif corriger les injustices sociales et construire de nouveaux critères d'appartenance à la communauté française. C'est pourquoi, madame la garde des sceaux, une réforme constitutionnelle moderne et ambitieuse se doit d'acter que le peuple s'exprime au pluriel et que, pour cette raison, le Parlement doit l'être aussi ! La parole est

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, dans ce débat sur l'évolution des droits du Parlement face au pouvoir exécutif, je partirai d'un constat assez clair en 2008, la majorité à laquelle j'appartenais, consciente de la nécessité de renforcer les droits du Parlement, et alors qu'on l'accusait de conforter « l'hyperprésidence », a approuvé la seule révision constitutionnelle de la V République à avoir renforcé significativement les droits des assemblées, à rebours de ce qui est envisagé aujourd'hui. Ainsi, elle a inscrit à l'article 24 de la Constitution la fonction de contrôle et d'évaluation du Parlement. Historiquement, avec le vote du budget, cette fonction de contrôle est la première à être apparue. Le Parlement, c'est d'abord une institution née de cette nécessité de contrôler le pouvoir. Nous pouvons être fiers de cette légitimité, de cette origine qui a fait du Parlement l'institution incarnant la liberté et la raison. Je sais que le Sénat y est profondément sensible. La révision constitutionnelle de juillet 2008, initiée par Nicolas Sarkozy, avait été précédée d'un riche débat, dont l'illustration la plus marquante est le travail du comité Balladur. Surtout, cette révision avait fait confiance au Parlement. Elle avait accepté de desserrer certaines sangles qui ne s'imposaient plus, en raison de la stabilité avec laquelle la VRépublique avait renoué. elle avait fait le choix de partager l'ordre du jour des assemblées et de renforcer le rôle des commissions parlementaires dans l'élaboration de la loi. En 2008, nous avons fait le pari de la maturité et de la responsabilité. Nous étions loin de ce climat de suspicion à l'égard de la représentation nationale. Nous avions conscience que, dans les rapports entre l'exécutif et le Parlement, une nouvelle étape devait s'ouvrir. Justement renforcer le Parlement, c'est aussi renforcer l'exécutif ; affaiblir le Parlement, c'est fragiliser l'exécutif, qui n'aura plus d'assise solide pour faire avancer ses réformes, et prendre le risque de le livrer aux aléas de la rue. Quand un sujet est grave pour la Nation, il vaut mieux qu'il soit débattu dans un hémicycle ! Rendre des comptes aux parlementaires, c'est un signe de démocratie, pas l'inverse. Quand l'exécutif est mieux contrôlé, il est en fait renforcé : il a davantage de légitimité pour décider, loin de tout sectarisme et de tout isolement. Les réformes du Parlement ne doivent pas être menées à l'insu des parlementaires. À cet égard, il faut faire confiance aux initiatives de nos assemblées, qui sauront trouver des instruments appropriés pour mieux contrôler l'exécutif. Le Sénat avait d'ailleurs fait preuve de créativité sur la question des droits du Parlement. Le débat d'initiative sénatoriale, institué en juin 2009, en est l'illustration. Notre assemblée a su être au rendez-vous quand il le fallait. Enfin, il y a un aspect foncièrement proche de la question des droits du Parlement : celui du nombre de parlementaires. Quand on envisage une réduction aussi sèche des élus de la Nation, en abrégeant les mandats en cours de la moitié du Sénat, ce qui ne s'est jamais vu dans les annales de la VRépublique, on risque d'affaiblir leurs missions, toutes leurs missions

Madame la garde des sceaux, comment peut-on envisager un contrôle efficace de l'exécutif, alors que vous souhaitez réduire si drastiquement le nombre de parlementaires et que vous envisagez de faire subir à certains élus une mesure d'exception indigne de notre démocratie ? Pourquoi ne pas, dans ce cas, raccourcir le mandat en cours du Président de la République ? La question du contrôle et celle du nombre de parlementaires sont, en réalité, coextensives : quand on affecte l'un, on affecte l'autre. Pour cette raison, nous serons vigilants dans les décisions que notre assemblée prendra en matière constitutionnelle et électorale. Nous refuserons ce couperet inique qui affaiblit les missions de notre assemblée. La parole

L'abstention, le rejet global du monde politique, la crise des formations partisanes traditionnelles, les votes extrêmes, des violences, parfois, dans l'expression des convictions politiques : autant d'éléments qui traduisent une réalité qu'on ne peut pas nier. Le vote de 2017, lors du scrutin présidentiel puis des élections législatives, a été clair : le besoin de rénovation est immense, et il serait illusoire de penser qu'on peut se dispenser d'y répondre avec une certaine force. J'insiste sur cet enjeu, car je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent considèrent que nos débats, finalement, ne les concernent pas et que nous serions engagés dans une discussion institutionnelle autocentrée. Au contraire, tout l'enjeu est pour nous de regagner la confiance de l'ensemble des Français.

Elle a été exposée par le Président de la République dans son discours au Congrès, le 3 juillet dernier. Le projet de loi constitutionnelle, dont vous avez bien voulu rappeler l'intitulé- « pour une démocratie plus représentative, responsable et efficace »

J'ai bien sûr entendu les interrogations et les critiques, mais aussi les soutiens à ces différentes propositions. Je partage avec vous vous la certitude que ces évolutions, dans leur ensemble, auront des conséquences sur la manière de concevoir la fonction parlementaire la fin du cumul des mandats a largement contribué à entamer cette évolution. Nous avons sans doute des pratiques différentes à imaginer, un nouveau type de relations à établir avec les citoyens

qui leur sont confiées par l'article 24 de notre Constitution : légiférer, contrôler l'action du Gouvernement et évaluer les politiques publiques. Mais rien de tout cela

Le projet de loi constitutionnelle entend tirer les conséquences des évolutions que notre pays a connues depuis la révision constitutionnelle de 2008, évolutions qui nous imposent de reconsidérer certains modes de fonctionnement de nos institutions, sans pour autant toucher à leur équilibre. Comme le Premier ministre l'a affirmé, cette révision constitutionnelle n'a pour objet ni un retour à la IVRépublique ni une aventure vers une VIRépublique. Il s'agit de respecter l'esprit des institutions, que le général de Gaulle, dans une célèbre conférence de presse de 1964, caractérisait par « la nécessité d'assurer aux pouvoirs publics l'efficacité, la stabilité et la responsabilité

une démocratie plus efficace, avec un Parlement qui légifère mieux- j'y reviendrai dans un instant -et évalue plus activement les lois et des collectivités territoriales qui peuvent répondre, par des capacités de différenciation et d'adaptation renforcées, aux demandes aux demandes concrètes des Français. Enfin, une démocratie plus responsable, avec un Parlement qui contrôle puissamment le Gouvernement et son administration, des ministres dont la responsabilité pénale relèvera désormais d'une juridiction de droit commun et une justice plus indépendante. Rien de tout cela ne traduit, pour reprendre les termes de Mme Assassi, un « coup de force », ni même une dérive autoritaire. Cette loi constitutionnelle n'est pas un verrou, monsieur Savoldelli, mais un élan !

de protéger le pouvoir exécutif. Bien des articles de notre Constitution s'expliquent à l'aune de cette volonté d'assurer une telle primauté

Le projet de révision constitutionnelle qui vous a été présenté voilà quelques jours n'inverse pas cette tendance. Il la conforte, tout en cherchant corrélativement à donner plus d'efficacité à l'action conduite tant par le Parlement que par le Gouvernement.

texte lui-même et éviter les procès d'intention. Je comprends, évidemment, la part de passion que soulèvent toujours les débats institutionnels, surtout lorsque ces débats sont menés par les premiers acteurs Je mesure bien les considérations politiques, jamais absentes des échanges d'arguments que nous aurons l'occasion d'avoir- et cela est bien naturel. Mais vous me permettrez, juste un instant, de revenir à des considérations très concrètes, qui figurent dans le texte proposé

et intitulé, montre bien que nous partageons une préoccupation, qui nous est commune. Le président du Sénat, dans son avant-propos, juge nécessaire de « rénover le travail parlementaire au service de la qualité de la loi et de la lutte contre l'inflation normative » et de « renforcer la fonction de contrôle et d'évaluation du Parlement au service d'une démocratie plus exigeante ». Nous ne disons pas autre chose ! Bien sûr, auront lieu sur les meilleures manières d'atteindre cet objectif. Le pouvoir constituant en débattra, mais l'essentiel, me semble-t-il, réside déjà dans ce diagnostic commun. Je suis d'ailleurs certaine que nos discussions seront de haute tenue, car je crois à la bonne foi de chacun, ainsi qu'à la conjonction des bonnes volontés. Je voudrais, à ce stade, souligner deux points essentiels à mes yeux la réforme institutionnelle que nous proposons n'entend ni remettre en cause le bicamérisme à la française ni porter atteinte aux droits du Parlement. Ce projet n'a nullement pour objet ou pour effet de remettre en cause le bicamérisme, tel qu'il a été voulu par le constituant de 1958.

Pour inégalitaire qu'il soit dans le texte même de la Constitution de 1958, le bicamérisme constitue l'un des piliers de notre régime constitutionnel, et nul ne songe à ébranler ces piliers.

De la sorte, nous proposons de renforcer au plan constitutionnel un mouvement que le Sénat a déjà engagé depuis 2015, sous l'impulsion du président Larcher, en cherchant à effectuer, de manière plus systématique, un contrôle des amendements les présidents de commission.

Il est simplement question de faire respecter les règles constitutionnelles. Qui pourrait soutenir qu'écarter des amendements de portée réglementaire ou sans incidence sur le fond du droit- je pense aux fameuses demandes de rapport qui fleurissent quasiment à chaque article de loi

le Gouvernement devra lui-même se soumettre à cette discipline rigoureuse, mais nécessaire pour atteindre l'objectif que nous partageons, celui d'une meilleure qualité de la loi. Toujours dans l'esprit de 2008, le projet s'inspire du dispositif que le Sénat a pérennisé dans son règlement de décembre dernier, en prévoyant, sur certains textes, la concentration des débats en séance publique sur les en séance publique sur les questions les plus essentielles, après un travail approfondi en commission. Cette meilleure articulation, également nécessaire, entre travail en commission

Après l'échec d'une CMP- c'est-à-dire quand les deux assemblées ont des positions irréconciliables -, et seulement dans ce cas, il est proposé de fusionner la nouvelle lecture et la lecture définitive à l'Assemblée nationale, selon une procédure plus resserrée.

à tirer les conséquences de la révision de 2008 et à répondre à la nécessité de désengorger l'ordre du jour de la séance. Le temps, le sénateur Bonhomme- le temps parlementaire, qui n'est pas nécessairement festonné des apparences du débat, pour reprendre vos propos -, est trop précieux

À cette fin, nous proposons une procédure prioritaire pour l'adoption de textes considérés par le Gouvernement comme particulièrement importants. L'idée est simple : l'ordre du jour, tel qu'il a été imaginé en 2008, est d'une rare complexité et soumet la navette parlementaire à une arythmie très préjudiciable au bon fonctionnement du Parlement. Le Sénat, en 2008, avait d'ailleurs relevé les problèmes qui pourraient naître de ce mécanisme complexe, et votre commission des lois, à l'époque, avait proposé un système plus simple. Le Gouvernement cherche une voie pour surmonter la difficulté. Ainsi que l'a montré le sénateur Alain Richard, dans tous les pays, on relève la force de l'exécutif pour préparer la loi,

S'il est indispensable de rendre plus fluide le travail législatif et, en quelque sorte, de le muscler, il est tout autant nécessaire- c'est une contrepartie

pèsent véritablement sur le cours des choses. Nous ne nous sommes pas approprié l'ensemble des moyens institutionnels à notre disposition, notamment en matière de contrôle.

et celui de la loi de règlement. Il s'agit, non pas de restreindre les droits du Parlement lors du débat initial, mais, au contraire, de conforter son pouvoir de contrôle au moment de l'examen de la loi de règlement. C'est à

puissent être inscrits à l'ordre du jour, sur l'initiative exclusive des assemblées. Je peine à voir en quoi une telle proposition réduirait les pouvoirs du Parlement. C'est, me semble-t-il, exactement le contraire ! Sans doute y a-t-il là, dans la certitude de la nécessité de ce contrôle effectif, quelque audace, quelque ambition, quelque modernité que M. le sénateur Savoldelli